monsieur le président,

Personnellement, je trouve que les retours en arrière ne font pas de bonnes politiques en avant, et que poursuivre les chimères ne mène à rien. La suppression de l'impôt sur la fortune, remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière- je le rappelle, celui-ci rapporte plus que prévu, nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'en parler a permis, je crois, en partie la baisse du chômage et l'une des meilleures croissances de l'Union européenne. [ ...] « On a besoin aujourd'hui que les gens qui possèdent de l'argent- pardonnez-moi le

pas encore pas tout à fait bien cadrée par la direction du budget ou par la direction de la sécurité sociale, mais il est prévu près de 6 milliards d'euros d'impôt sur le revenu en moins par rapport au PLF présenté en décembre dernier et environ 4,5 milliards d'euros

de nos échanges politiques dans le cadre de la loi de finances, mais aussi sur d'autres sujets, il existe deux lignes de partage, des stratégies et des explications différentes. Pour notre part, nous pensons que nous sommes depuis assez longtemps dans un cycle politique,

Pourtant, à l'époque, on n'entrait pas dans la crise, on commençait, en tous les cas on l'espérait, à pouvoir en sortir. Mais souvenez-vous de ce que vous avez fait cette année-là. Sur les mêmes arguments,

d'euros. Que s'est-il passé dix-huit mois plus tard, en décembre 2013, lors des voeux du Président de la République au Français : machine arrière toute ! Si, pendant les dix dernières années- je veux bien exclure la période 2007 -, si, pendant le quinquennat de François Hollande, nous n'avons pas réussi à relancer la croissance ni à inverser la courbe du chômage et de la dette, c'est certainement parce que, à l'été 2012, vous vous êtes trompés

monsieur le ministre

conflit commercial avec les États-Unis lié à la fameuse taxe Trump, incertitudes autour du Brexit, instabilité des marchés internationaux, notamment asiatiques ... Et pourtant, les dépenses nécessitées par les travaux de la vigne courent La viticulture française traverse aujourd'hui une grave crise, dont une partie du secteur ne se relèvera pas. Cette crise, qui frappe d'abord les professionnels, inquiète sérieusement les élus des terroirs viticoles que nous représentons. Dans

La survie des acteurs de la vigne et du vin est essentielle à la bonne santé économique de ces territoires. Pour de nombreux vignerons, la fermeture des restaurants, cafés et bars, auprès desquels ils écoulaient une partie de leur production, entraîne des conséquences Les viticulteurs comptent beaucoup sur leur réouverture, d'autant que les achats dans la grande distribution ont fortement chuté. Pour accompagner la réouverture des cafés et restaurants et embarquer la filière viticole dans une reprise d'activité tant espérée, je propose d'aligner le taux de TVA appliqué aux aux produits d'origine viticole, dont le vin est le représentant emblématique, sur celui des autres produits servis dans la restauration. Aujourd'hui, les vins et eaux-de-vie de vin se voient appliquer un taux de 20 %, alors que les boissons non alcoolisées et les autres produits servis en restauration bénéficient d'un taux de 10 % ou de 5,5 %.

Monsieur le ministre, sur cet amendement,

à instaurer une taxe due par les services de communication des moteurs de recherche comme Google au profit des publications de presse, au titre de l'exploitation qui est faite de leurs articles et de leurs référencements. Cette taxe, qui a vocation être temporaire, vise à mettre en application de toute urgence les dispositions de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse durant les négociations entre les plateformes et les éditeurs En effet, si la loi est maintenant promulguée depuis plus de six mois, les premières estimations montrent qu'il faudra attendre encore un an au moins avant qu'elle ne soit pleinement appliquée. Au regard de la fragilité économique du secteur de la presse, cette période pourrait être fatale à certains titres. Il est donc urgent d'agir selon monsieur le rapporteur général,

Afin d'accompagner les collectivités territoriales qui doivent faire face à la crise du Covid-19, cet amendement vise à inclure dans le champ du FCTVA les achats de protections individuelles telles que les masques, blouses, gels hydroalcooliques par les collectivités territoriales à destination des professionnels de santé dans un premier temps et, plus tard, de leurs administrés.

le Premier ministre, le pôle collectivités locales et le pôle Bercy, en l'occurrence Olivier Dussopt et moi-même, consultons beaucoup les collectivités locales pour connaître précisément

117 millions !-, alors qu'il en fallait au moins 30 à 40 millions par semaine pour le seul personnel soignant.

du carburant va diminuer, mais vous savez très bien, mes chers collègues, que, compte tenu des taxes que supporte le carburant, la diminution du prix à la pompe n'est absolument pas proportionnelle à la chute du prix du baril de pétrole.

consécutive à la revalorisation de l'engagement local, notamment dans le cadre de la loi Engagement et proximité. Il s'agit de faire entrer 3 500 communes rurales de moins de 500 habitants dans ce dispositif.

Beaucoup d'entre vous doivent se dire que leur commune n'aura pas les moyens de financer cette remise à niveau de leur indemnité. Nous allons donc proposer un effort ciblé, mais substantiel, sur la dotation particulière pour les élus locaux : nous proposerons de la doubler pour les communes éligibles de moins de 200 habitants et de l'augmenter de 50 % pour les communes éligibles de 200 à 500 habitants. C'est une façon de garantir le fait que les mesures qui ont été proposées peuvent entrer en vigueur de façon pérenne pour ceux qui sont concernés. » » Aujourd'hui, les communes concernées s'aperçoivent que leur DPEL n'a pas été augmentée comme cela leur avait été promis et qu'un critère supplémentaire de potentiel fiscal a été introduit pour réduire le coût de la mesure. mesure. À l'heure où le Président de la République en appelle aux maires pour mener à bien le déconfinement, il manque 8 millions d'euros pour honorer cette promesse.

Monsieur le ministre,

300 et 400 millions d'euros par mois, soit entre 600 et 800 millions d'euros pour les seuls mois de mars et d'avril. Leurs provisions vont donc être bien supérieures aux résultats de l'assurance dommage, ce qui justifie d'affecter les recettes ainsi dégagées au soutien des

Aujourd'hui, mes chers collègues, je vous le dis : les assurances doivent être au rendez-vous de la mobilisation économique.

sanitaire, un certain nombre d'activités économiques ont été interdites. On a donc déplacé la marge, puisque l'on a créé, pour certains secteurs, une rente par décision administrative. C'est la loi classique de la concurrence, du monopole, etc. Bref, on a déplacé la rente. Il n'est donc pas illogique

les assureurs traînent un peu les pieds. Il faut leur mettre la pression, et nous sommes à vos côtés pour cela

à Mme Jocelyne Guidez. Le présent amendement vise à rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l'assurance, mise en place en 2011 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. L'économie française, durement affectée par la crise sanitaire sans précédent générée par l'épidémie de Covid-19, doit être aujourd'hui massivement soutenue par les acteurs de l'assurance, bénéficiaires malgré eux de la chute significative du nombre de sinistres couverts. Le produit de ladite taxe devra être mis à profit pour soutenir les actions en faveur des TPE et PME. Les deux

pour bénéficier d'un contrat assez large du point de vue assurantiel. Aujourd'hui, ils enregistrent tous des pertes d'exploitation, et ils se retrouvent sur le carreau,

compte tenu des nécessaires réserves prudentielles. J'ai entendu ce qu'a dit à l'instant M. le ministre sur les discussions avec le secteur de l'assurance. J'ai également entendu ce qu'a dit Bruno Retailleau, et je le suivrai volontiers dans son argumentation. Nous aurons dans

des assurances sont transparents. Pour les assurances de biens, en 2018, la Fédération française de l'assurance signale 56 milliards d'euros de cotisations,

qui paye ses cotisations d'assurance parce que c'est un honnête homme, mais qui a interdiction de vendre ses produits. Je pense à un ami kinésithérapeute, qui s'est installé il n'y a pas longtemps. En plus

auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit ... Le montant du prélèvement serait fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1 avril